La séance est ouverte. Le compte rendu intégral de la séance du mercredi 17 janvier 2018 a été publié sur le site internet du Sénat. Il n'y a pas d'observation ? ... Le procès-verbal est adopté.

L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social

Lors des questions d'actualité au Gouvernement de la semaine dernière, deux sénateurs ont interpellé le Premier ministre à propos de différentes démarches qui, initiées par le ministère de la recherche et plusieurs universités, nous semblaient constituer des transpositions anticipées du projet de loi relatif à l'orientation et à la réussite des étudiants

Toujours la semaine dernière, le samedi 20 janvier, a été publié au un arrêté ministériel destiné à préciser le fonctionnement de la plateforme « Parcoursup » dans le cadre de la procédure nationale de préinscription, qui constitue l'une des dispositions essentielles de la loi que nous aurons à examiner. Il est très regrettable qu'aucune information sur cet arrêté ministériel n'ait été donnée par la ministre à notre commission lors de son audition. Sur le fond, il nous semble très contestable de publier ainsi un arrêté découlant de l'application d'une loi qui n'a pas encore été votée par notre Haute Assemblée. Enfin, cette anticipation très discutable fait peser sur les familles des risques de contentieux juridiques importants, alors qu'il leur est demandé de commencer, dès cette semaine, à introduire leurs voeux sur ce nouveau portail. À tout le moins, nous souhaiterions que soit rappelée au Gouvernement par notre Haute Assemblée la règle constitutionnelle, simple, selon laquelle une loi ne peut être appliquée qu'après son adoption définitive et sa promulgation. Nous nous réservons le droit de déférer cet arrêté devant la juridiction administrative. Acte vous est

Monsieur le président, monsieur le rapporteur- cher Alain Milon -, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, « ce n'est pas dans l'objet que réside le sens des choses, mais dans la démarche », écrivait Antoine de Saint-Exupéry. En effet, c'est bien tout au long de leur processus de maturation, par lequel nos projets communs, en se nourrissant des aspirations et des apports de chacun, se concrétisent, qu'ils puisent leur sens profond et leur force. Cette affirmation illustre la nature même du débat parlementaire comme la philosophie générale de la réforme qui nous réunit à nouveau aujourd'hui, celle du renforcement du dialogue social. Cette réforme, qui, par son processus d'élaboration, son ampleur et sa visée,

au terrain ; d'autre part, son corollaire, la responsabilisation des acteurs, qui doivent se mobiliser et s'emparer des opportunités offertes pour relever les défis présents et à venir. C'est pourquoi cette réforme, qui est essentielle pour la réussite de la transformation de notre modèle social, a été portée par une démarche pragmatique et dynamique et s'est matérialisée par les ordonnances, adoptées à la suite de la loi d'habilitation que vous avez votée. Annoncées pendant la campagne présidentielle, ces ordonnances sont le fruit, vous le savez, d'une coconstruction inédite, alliant démocratie sociale- plus de 300 heures de discussions -et démocratie politique.

que cette loi soit promulguée dès le 15 septembre dernier. Le mandat de la loi d'habilitation que vous avez votée était clair : il s'agissait de prendre, dans les meilleurs délais, les mesures nécessaires pour créer les conditions d'un dialogue social structuré, lisible, décentralisé offrant plus d'agilité et de sécurité tant aux employeurs qu'aux salariés et à leurs représentants, qui seront, dans ce cadre équilibré, des acteurs responsabilisés, plus formés et mieux armés pour envisager cette négociation, et l'avenir Comme nous nous y étions engagés, nous avons appliqué ce mandat sans attendre. Ainsi, sept jours après la promulgation de la loi d'habilitation, soit le 22 septembre dernier, cinq ordonnances ont été publiées au, ce qui a permis l'entrée en vigueur immédiate d'une grande partie des dispositions.

peuvent d'ores et déjà s'emparer des opportunités permises par les ordonnances pour libérer les initiatives, protéger chacun et dynamiser l'emploi. C'est ce mouvement de confiance et de responsabilisation qu'ont amplifié vos collègues députés,

D'ailleurs, en sillonnant la France depuis la publication des ordonnances, j'ai pu constater- comme vous, je le pense -l'effet psychologique réel produit par les ordonnances, en particulier dans les petites et moyennes entreprises. Nous avons éteint une peur et redonné confiance aux chefs d'entreprise pour embaucher, au moment même où les carnets de commandes se remplissent et où la croissance repart avec robustesse. La confiance en l'avenir est essentielle pour transformer ces possibilités en embauches Ce changement tient d'abord au fait que les ordonnances transforment, à travers le droit, l'esprit même du code du travail comme du dialogue social, qui est renforcé.

Comme vous le savez, cette nouvelle articulation entre la loi, l'accord de branche et l'accord d'entreprise repose sur un système supplétif qui constitue un filet de sécurité pragmatique faute d'accord d'entreprise, c'est l'accord de branche qui s'applique ; faute d'accord de branche, c'est la loi. Et, dans certains domaines, comme les salaires hiérarchiques, les grilles de classification, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ou la prévoyance, l'accord de branche s'impose aux entreprises. Il existe donc un véritable équilibre entre les accords d'entreprise, les accords de branche et les principes fixés dans la loi. En outre, la branche professionnelle a un pouvoir de verrou, en décidant qu'un accord d'entreprise devra respecter au minimum ses stipulations, et ce dans quatre domaines. Le premier domaine concerne la gestion et la qualité de l'emploi.

Un rôle central est ainsi dévolu à la négociation de branche, dont l'insuffisance actuelle explique, en partie, pourquoi les entreprises n'emploient toujours que 3,3 % de salariés handicapés, alors que, depuis plus de vingt ans, l'objectif est d'atteindre 6 %. Il est temps de convenir que nous sommes tous responsables de cette situation. Les mécanismes prévus par la loi doivent pousser à la négociation de branche qui, elle seule, nous permettra de progresser significativement.

soit avec un élu du personnel, soit avec les salariés dans les entreprises de moins de 20 salariés qui n'ont pas d'élu du personnel. Ce nouveau système de consultation permettra d'éviter une procédure lourde, tout en garantissant aux salariés une autonomie de jugement et d'appréciation et une liberté de parole, puisqu'il faut que deux tiers d'entre eux soient d'accord et que leurs délibérations se tiennent hors de la présence du chef d'entreprise. Il est clair que ce dialogue informel existe dans de très nombreuses petites et moyennes entreprises, de manière très positive, mais il est désormais sécurisé là où il existait et encouragé là où il n'était pas pratiqué. Pour les entreprises de plus de 50 salariés, le dialogue social est également simplifié et amplifié et rendu plus opérationnel par la fusion des trois instances d'information et de consultation en une seule

que les compétences du délégué du personnel, du comité d'entreprise et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Je tiens à souligner que les entreprises pourront se doter,

Comme vous le savez, une étape supérieure peut être franchie, par accord majoritaire, pour mettre en place un conseil d'entreprise qui intègre l'ensemble des fonctions de représentation du personnel- information, consultation, mais aussi négociation par l'intermédiaire des délégués syndicaux.

L'extension des champs de négociation ouverts contribuera à ce phénomène, mais cette capacité d'anticiper et de s'adapter rapidement aux évolutions du marché ne sera accessible que si les entreprises arrivent à conclure des accords majoritaires sur le temps de travail, la rémunération ou la mobilité.

Cette agilité par le dialogue social, qui permet d'anticiper, d'accompagner, de moderniser, d'augmenter la performance économique et de favoriser le progrès social, s'inscrit dans un cadre juridique équilibré, à même de libérer

d'iniquité. Comme nous nous y étions engagés, les ordonnances lèvent ces barrières par le biais de plusieurs mesures de simplification et de clarification pour davantage de transparence et d'équité.

ce code sera adapté. Ce dispositif est significatif de notre volonté commune de rendre effectifs les droits des salariés dans leur vie professionnelle au quotidien. Nous avons aussi pris le parti de l'audace, en établissant, c'est une première en Europe, un droit au télétravail sécurisé et souple. Il s'agit d'un droit opposable, auquel le salarié peut demander à bénéficier ; il appartiendra à l'employeur de proposer une négociation aux partenaires sociaux, d'élaborer une charte et de se justifier s'il ne peut donner suite à la demande. Nous pensons qu'il s'agit d'une évolution de société importante, qui peut permettre

et nous avons trouvé une formule opérationnelle et pragmatique pour que ce droit ne soit pas seulement formel, mais qu'il puisse être exercé dans toutes les entreprises. Désormais, pour les trois critères ergonomiques, un examen médical permettra de mettre en évidence les conséquences de conditions de travail pénibles et le salarié pourra partir deux ans plus tôt à la retraite à taux plein.

Les conclusions de cette mission nous seront remises en février 2018. En complément, nous avons chargé la députée Charlotte Lecocq, l'ancien secrétaire confédéral syndical Henri Forest et la personnalité qualifiée Bruno Dupuis

Enfin, pour en revenir au mandat que vous nous avez délivré, nous avons sécurisé davantage les relations de travail, notamment au moment de leur rupture. Ainsi, concernant le licenciement, les ordonnances mettent un terme à la prévalence du vice de forme sur l'examen au fond par le juge- c'est un point essentiel.

par l'affichage des emplois disponibles ou grâce à l'intranet de l'entreprise. Elles harmonisent à un an les délais de recours en cas de contestation de la rupture du contrat de travail. S'agissant des indemnités légales de licenciement, nous avons respecté l'engagement pris devant la représentation nationale. Nous les avons augmentées de 25 %. Je rappelle qu'auparavant un salarié gagnant 2 000 euros percevait 4 000 euros d'indemnités après dix ans d'ancienneté ; il en percevra désormais 5 000. Quant aux indemnités prud'homales, les ordonnances instaurent, comme annoncé, un barème de dommages et intérêts reposant sur plancher et un plafond, ce qui sécurise les deux parties, en donnant plus de visibilité sur les contentieux potentiels, et incite à la conciliation. Je rappelle que, comme je m'y étais engagée, le plafond ne s'applique pas en cas d'atteinte aux libertés fondamentales, de harcèlement ou de discrimination. L'actualité de ces deniers mois l'a montré avec le harcèlement, il s'agit non pas simplement d'une perte d'emploi, mais bien d'une atteinte à l'intégrité de la personne. C'est pour cela que, dans ces situations, le plafond ne s'applique pas. L'incitation à la conciliation se manifeste également par l'instauration de la rupture conventionnelle collective, qui transpose au niveau collectif ce qui a fonctionné au bénéfice des deux parties de manière individuelle. Cette rupture conventionnelle collective ne vise pas toutes les situations, elle permet à une entreprise qui souhaite se réorganiser, anticiper, se restructurer,

Accorder plus de grain à moudre au dialogue social nécessite de donner les moyens aux différents partenaires d'en être pleinement acteurs. Or, aujourd'hui les vocations syndicales sont insuffisantes par crainte, pour les élus, de s'enfermer dans leur mandat. Il faut donc renforcer l'attractivité du mandat syndical. C'est le sens de la mission que j'avais confiée à Jean-Dominique Simonpoli, directeur général de l'association Dialogues, qu'il poursuit désormais avec Gilles Gateau, directeur général des ressources humaines d'Air France.

qui existe dans les faits, comme l'a montré un rapport du Conseil économique social et environnemental. C'est pourquoi je ne peux qu'exprimer le regret que vous ayez supprimé cet outil en commission. Enfin, conformément aux engagements du Président de la République, nous évaluerons, de façon transparente et efficace, avec les partenaires sociaux et le Parlement les effets de cette loi. J'ai en ce sens confié une mission à Sandrine Cazes, de l'OCDE, ainsi qu'à Jean-François Pilliard et Marcel Grignard-

le passé nous retient, c'est pour ça que le présent nous échappe ». Prouvons-lui, par la ratification de cette première réforme structurelle, qu'il avait tort ! L'avenir ne nous tourmente pas, le passé ne nous retient pas et le présent ne nous échappe pas ! Il est aujourd'hui entre vos mains. Donnons à nos concitoyens l'audace et la capacité d'être pleinement acteurs de leur vie professionnelle et de construire

sociales, rapporteur. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nous examinons aujourd'hui l'une des plus importantes réformes du droit du travail menées ces trente dernières années, qui devrait redonner confiance à nos concitoyens dans la capacité de notre pays à se moderniser et à restaurer sa compétitivité. L'habilitation donnée par le Parlement au Gouvernement, au mois d'août dernier, pour procéder par ordonnances au renforcement du dialogue social visait quatre objectifs principaux : donner une place centrale à la négociation d'entreprise, mieux assurer la représentation du personnel, sécuriser les licenciements et adapter les règles de prévention des risques professionnels. Le Sénat avait imprimé sa marque sur la loi d'habilitation, notamment en autorisant les employeurs à organiser un référendum pour valider un projet d'accord collectif, en garantissant la transparence des comptes de la nouvelle instance unique de représentation du personnel, ou encore en imposant un périmètre national pour apprécier la cause économique d'un licenciement quand l'entreprise appartient à un groupe. Moins de trois mois après le dépôt du projet de loi d'habilitation à l'Assemblée nationale, le Gouvernement a adopté, le 22 septembre 2017, cinq ordonnances denses et techniques qui traduisent ces orientations, à l'issue d'une concertation atypique, mais approfondie, avec les partenaires sociaux. Les députés ont adopté, le 28 novembre dernier, le projet de loi de ratification, assorti d'une cinquantaine d'amendements n'ayant pas dénaturé l'équilibre général des ordonnances. La plupart d'entre eux ont ont apporté des précisions pertinentes, ont corrigé des imperfections, inévitables en raison de l'ampleur du chantier et des délais imposés aux services du ministère, ou ont enrichi les dispositifs, par exemple en relevant la limite d'âge pour les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Il appartient désormais au Sénat de se prononcer sur la ratification des ordonnances afin de leur donner valeur législative. Lors de l'examen du projet de loi de ratification, le 20 décembre dernier, la commission des affaires sociales a résolument approuvé la philosophie des ordonnances, qui s'inscrivent dans une tendance de fond trouvant son origine dans la position commune du 16 juillet 2001, au travers de laquelle les partenaires sociaux appelaient à développer la négociation collective. Cet appel a trouvé sa traduction dans plusieurs textes, comme la loi du 4 mai 2004, qui a permis aux accords d'entreprise de déroger aux accords de branche, ou, plus récemment, la loi Travail du 8 août 2016, qui a donné la primauté à l'accord d'entreprise sur l'accord de branche pour fixer les règles en matière de durée du travail, de congés et de repos. Surtout, ces ordonnances reprennent et approfondissent des propositions défendues de manière constante par la majorité sénatoriale depuis 2014. Je pense notamment à la simplification des accords de flexisécurité, à la modulation dans le temps des effets des décisions du juge, à la suppression des contrats de génération, à la rationalisation des institutions des institutions représentatives du personnel, ou encore à la simplification du compte personnel de prévention de la pénibilité. L'ensemble de ces mesures contribue à répondre aux difficultés auxquelles chacun d'entre nous a été sensibilisé, dans son département, au contact des acteurs économiques. Dès lors, nos travaux ont été guidés par quatre principes, qui avaient déjà servi de fil conducteur au Sénat lors de l'examen du projet de loi d'habilitation la simplification des normes, le renforcement de la compétitivité de l'économie, la prise en compte des spécificités des petites entreprises et la protection des droits fondamentaux des salariés. la commission a adopté trente-sept amendements, dont trente-six sur mon initiative. Si certains d'entre eux tendaient à corriger des erreurs de rédaction ou des malfaçons, d'autres visaient à revenir sur certains choix du Gouvernement. Le Parlement a toute latitude pour modifier le présent projet de loi, quitte à priver de base légale les textes réglementaires d'application des ordonnances, qui ont tous déjà été publiés, ou à les modifier. Depuis nos travaux communs sur la loi d'habilitation, j'ai établi une relation de confiance avec Mme la ministre et son cabinet, ce dont je me félicite. Pour autant, je suis en désaccord avec certains des arbitrages rendus, qui, sur plusieurs points, ne correspondent pas à la position constante de notre assemblée, ou qui, sur d'autres, me sont apparus trop éloignés de l'habilitation que nous avons conférée Nous les avons donc modifiés, et j'espère pouvoir convaincre le Gouvernement, ainsi que nos homologues de l'Assemblée nationale, du bien-fondé de la position du Sénat d'ici à la commission mixte paritaire. Ainsi, pour favoriser la négociation collective, nous avons approuvé la création d'un accord unique et simplifié de flexisécurité, que nous avons baptisé « accord de performance sociale et économique ». Les leçons des échecs précédents en la matière semblent avoir été tirées, bien que le volet relatif à l'accompagnement des salariés licenciés à la suite de leur refus d'appliquer un tel accord mériterait, à mes yeux, d'être amélioré. De plus, nous avons facilité la conclusion d'accords collectifs avec les représentants élus du personnel dans les entreprises dépourvues de délégué syndical. Enfin, fidèles à la position exprimée par le Sénat depuis 2016, nous avons supprimé l'accélération de la généralisation des accords majoritaires, considérant que la date du 1 mai 2018 retenue dans l'ordonnance pourrait freiner la conclusion d'accords d'entreprise. La commission a également approuvé la fusion des institutions représentatives du personnel au sein d'une structure unique, le comité social et économique, le CSE. Il lui a toutefois semblé important de renforcer les obligations de celui-ci en matière de transparence financière, obligations qui s'appliquent déjà depuis quatre ans aux comités d'entreprise grâce à la persévérance de notre collègue Catherine Procaccia. Nous avons ainsi souhaité que tous les CSE qui remplissent au moins deux des trois critères suivants- employer au moins 50 salariés, avoir des ressources dépassant 3,1 millions d'euros, disposer de plus de 1,55 million d'euros de patrimoine -soient dotés d'une commission des marchés, chargée de fixer des critères objectifs pour choisir ses prestataires. Les partenaires sociaux de l'entreprise ne pourront plus convenir, par accord, de s'en dispenser. De même, nous avons rendu obligatoire la formation de tous les membres du CSE aux problématiques de santé et de sécurité au travail, formation qui pouvait être restreinte aux membres de la commission dédiée, car c'est l'instance elle-même qui reste compétente pour rendre un avis à l'employeur sur ces sujets. Soucieuse de sécuriser les relations de travail, la commission a fixé à trois mois le délai dont dispose le juge pour se prononcer en cas de recours en nullité contre un accord collectif ou de contestation d'un avis du médecin du travail. Elle a précisé que toute fraude rendait caduque l'utilisation d'un périmètre national pour apprécier, au sein d'un groupe, la cause économique d'un licenciement. En outre, s'agissant de la rupture conventionnelle collective, elle a autorisé les entreprises dépourvues de CSE à y recourir et a précisé que l'administration, quand elle examine le volet relatif à l'accompagnement et au reclassement des salariés qui acceptent cette rupture, devait seulement exercer un contrôle minimum, et non d'opportunité. Enfin, nous avons veillé à ce que les ordonnances n'outrepassent pas le champ des habilitations. C'est pourquoi nous avons refusé toute dérogation à l'interdiction d'effectuer plus de trois mandats consécutifs de représentation du personnel, sauf dans les entreprises de moins de 50 salariés.

aux partenaires sociaux de se saisir des nombreuses souplesses qu'elle leur offre, et au Gouvernement de les accompagner en ce sens. Au vu des enjeux, je ne doute pas qu'ils se mobiliseront dès maintenant afin de remporter la bataille de l'emploi et de restaurer la compétitivité de l'économie française. Il va sans dire que le Parlement se montrera très attentif, dans les mois à venir, à l'évaluation de ces dispositions, mais également à la stabilité de ce nouveau cadre juridique : c'est à ce prix que l'atmosphère de confiance actuelle pourra être pérennisée. Nous passons Nous passons à la discussion de la motion tendant à opposer la question préalable.

: il s'agit d'éviter que l'on aborde le fond de votre projet, à savoir la poursuite et l'amplification de la démolition du code du travail. La mise en scène très théâtralisée de la signature de ces ordonnances par le président Macron ne leur confère pas, pour autant, un caractère plus populaire. Ainsi donc, le Gouvernement a décidé de contourner le Parlement en démultipliant le recours aux ordonnances. Aujourd'hui, les ordonnances sont utilisées pour réformer le code du travail, mais, demain, le Gouvernement a l'intention d'y avoir recours pour mettre à mal les centres de santé en les transformant en centres lucratifs, pour réformer le logement social ou encore le secteur agricole, à la suite des états généraux de l'alimentation, cette liste n'étant pas exhaustive. Le Gouvernement souhaite passer en force sur des sujets aussi importants ; nous nous y opposons, car, pour nous, madame la ministre, cela remet en cause le contrôle par la représentation du peuple. Ce caractère antidémocratique se ressent bien évidemment jusque dans notre assemblée, puisque notre pouvoir d'intervention est plus que restreint. Le principe des ordonnances est l'octroi d'un blanc-seing au Gouvernement, ce qui remet profondément et dangereusement en cause notre droit d'élaboration de la loi. De plus, mes chers collègues, en toute honnêteté, lequel d'entre nous peut prétendre maîtriser à 100 % le contenu très technique de ces cinq ordonnances ? C'est, je le redis avec gravité, un vrai problème démocratique que de ratifier un texte dont on ne maîtrise pas totalement les tenants et les aboutissants et que l'on

Votre rapporteur considère que le recours aux ordonnances, s'il est prévu par la Constitution, ne permet pas en l'espèce la tenue d'un débat satisfaisant au Parlement, compte tenu notamment de l'ampleur des thèmes traités. venons-en au fond. La réduction des droits collectifs des salariés est le premier grand chantier de votre quinquennat. Cela s'inscrit, hélas, dans le droit fil de l'action du gouvernement précédent, au nom d'une prétendue modernisation du code du travail.

Peu importent les résultats en matière d'emploi, finalement, tant que les grands patrons peuvent engranger plus de profits et licencier avec plus de souplesse. Nous l'avons rappelé lors des débats sur le projet de loi d'habilitation, en juillet dernier

C'est également vrai à l'échelle européenne avec les « minijobs » à l'allemande, les contrats « zéro heure » à l'anglaise, le à l'italienne ou encore les « reçus verts », comme au Portugal. ont peut-être permis de dégonfler artificiellement les statistiques du chômage, mais ils ont précarisé les travailleuses et les travailleurs en plongeant nombre d'entre elles et eux dans la misère, sans produire aucun effet réel et durable sur l'emploi. on nous reproche souvent, à nous parlementaires communistes, d'être caricaturaux, voire binaires, mais, malheureusement, nous ne décrivons que des faits bien réels, que tout un chacun peut vérifier. Les salariés de notre pays vivent de plus en plus mal et se rendent compte quotidiennement de la précarisation de leur emploi. Ils sont aussi conscients que les instances représentatives du personnel, les IRP, qui étaient là, avec les syndicats, pour les défendre, les protéger, sont, elles aussi, attaquées,

Les justifications que vous avancez -les syndicats ne sont pas présents partout, le taux de syndicalisation recule, il faut redonner la parole aux salariés -ne tiennent pas à l'épreuve de la réalité des rapports de force dans les entreprises. Sans entrer dans le détail des ordonnances, car mon collègue Dominique Watrin le fera tout à l'heure si cette motion est rejetée- mais on peut toujours rêver à son adoption, surtout en cette période des voeux ! -, je veux redire ici que les principales mesures que le Gouvernement est en train de mettre en oeuvre vont conduire à un véritable dumping social. Vous êtes en train de créer une société de l'individualisation, où tout se négociera, rien ne sera plus garanti : primes d'ancienneté, de panier, de nuit, pour ne citer que quelques exemples, ne seront plus sanctuarisées. Sur tous les sujets qui ne seront pas mentionnés explicitement dans le code du travail, l'accord d'entreprise prévaudra sur l'accord de branche, même lorsqu'il est moins favorable aux salariés niveau de prise en charge des arrêts maladie au-delà des minima sociaux, congés exceptionnels pour événement familial, pour enfant malade ou maternité au-delà des minima légaux. Ce sont autant de remises en cause de droits conquis, qui vont affecter négativement les conditions de travail de tous les salariés, et singulièrement des femmes. De plus, vous supprimez l'une des rares avancées à mettre au crédit du précédent gouvernement, à savoir le compte de prévention de la pénibilité. Vous prétendez vouloir renforcer le dialogue social, comme l'indique l'intitulé du projet de loi, permettre à l'échelon le plus local, à savoir l'entreprise, de définir ce qui est bon pour lui, mais c'est nier totalement, nous n'avons eu de cesse de le répéter, le rapport de force, le lien de subordination, la hiérarchie qui existent au sein de toute entreprise, pour tout contrat de travail. La loi est justement là pour protéger, fixer un cadre général, éviter les abus. Avec votre réforme, vous abrogez purement et simplement les principes fondamentaux de notre code du travail. Au lieu de l'égalité devant les droits, inscrite dans notre Constitution, vous mettez en place une variabilité des droits, une inégalité entre les salariés. Pourtant, vous continuez à assurer que les salariés seront mieux protégés grâce à vous, que leurs conditions de travail s'amélioreront. Comment, dès lors, expliquer que le MEDEF soit si satisfait de votre beau projet et que votre texte ait été largement soutenu par la majorité à l'Assemblée nationale, comme il va l'être également par la majorité sénatoriale ?

de débat orchestré par le Gouvernement. Ainsi, certaines ordonnances sont déjà entrées en application, sans l'aval du Parlement. Dès lors, à quoi bon débattre ? Même si le Parlement ne les ratifiait pas, les ordonnances s'appliqueraient sous forme réglementaire.

Vous consultez pour la forme, puis vous agissez comme prévu : drôle de conception du dialogue social ! De même, madame la ministre, vous vous êtes vantée d'avoir rencontré, depuis la publication des ordonnances, plus de 3 000 chefs d'entreprise, et, avec votre équipe, plus de 5 000 directeurs des ressources humaines, ce qui vous aurait permis de constater l'effet psychologique réel produit par les ordonnances sur les PME. C'est une bonne chose

mais nous ne sommes pas maîtres du règlement du Sénat. Je rappellerai enfin à celles et ceux qui nous reprochent de recourir à la motion tendant à opposer la question préalable que la majorité sénatoriale l'a utilisée lors de l'examen du projet de loi de finances rectificative pour 2017 et lors de la seconde lecture du PLFSS pour Parce que le Gouvernement a, en réalité, refusé le débat sur ces ordonnances, parce que le Gouvernement affirme que l'égalité entre les femmes et les hommes sera une priorité du quinquennat, mais supprime les CHSCT au moment même où des milliers de femmes dénoncent le harcèlement sexuel, notamment sur leur lieu de travail,

tendant à opposer la question préalable, car je considère que, sur la forme, le recours aux ordonnances est justifié quand il faut agir rapidement sur des sujets techniques. J'ajoute que le Parlement n'est pas totalement dessaisi de ses prérogatives en cas de recours aux ordonnances, car c'est lui qui fixe le champ de l'habilitation, qui doit être précis, et le délai pour déposer le texte de ratification. lorsqu'il examine, comme nous le faisons aujourd'hui, le projet de loi de ratification, il peut approuver les dispositions des ordonnances, les modifier, voire les supprimer. Ce pouvoir du Parlement n'est pas remis en cause par la publication des textes réglementaires d'application. Sur le contenu des ordonnances, je dirai simplement qu'elles donnent une place

que nous sommes aujourd'hui appelés à approuver. Afin que le projet de loi fasse l'objet d'un vrai débat, l'Assemblée nationale a souhaité le réorganiser pour que chaque segment de la réforme mise en oeuvre au travers de ces ordonnances puisse être pleinement discuté. Je souhaite préciser la position du groupe Les Indépendants-République et Territoires sur les grandes orientations de ces ordonnances. Le Gouvernement a d'abord défini le principe de la primauté de l'accord d'entreprise, afin de faciliter la négociation collective dans toutes les entreprises, plus particulièrement dans les plus petites C'est la première fois qu'une réforme du code du travail donne la priorité aux TPE et PME. Cela mérite d'être souligné. Elles pourront désormais conclure un accord collectif, même en l'absence de délégué syndical. Il faut savoir que 4 % seulement des PME disposent d'un délégué syndical. Cette simplification de la vie quotidienne des TPE et PME passe par une série de mesures attendues de longue date : réforme des règles de licenciement, nouveau barème des dommages et intérêts et suppression des contraintes administratives inapplicables, notamment. Ces ordonnances clarifient les règles, tout en favorisant l'instauration d'un climat serein entre le chef d'entreprise et les salariés. Elles nous semblent susceptibles de redonner confiance en donnant les moyens d'anticiper et de s'adapter aux nouvelles contraintes de la vie économique et financière. Pour atteindre ces objectifs, le Gouvernement a proposé la fusion des instances d'information et de consultation en une nouvelle structure, le conseil social et économique. Simplicité, efficacité, rapidité : tels sont les mots d'ordre. Je ne reviendrai pas dans le détail sur toutes les mesures figurant dans ces textes, mais je souhaite insister sur le fait que, si elles visent à aider les entreprises à relever les défis de l'économie du XXI siècle, elles ouvrent aussi de nouveaux droits pour les salariés et consacrent de nouvelles garanties pour les syndicats et les élus du personnel.

Bien sûr, ces ordonnances peuvent être complétées. Notre collègue Daniel Chasseing fera part des propositions de notre groupe sur ce point. ces ordonnances ne sont qu'une pierre d'un vaste édifice. Cette réforme du dialogue social devra s'accompagner d'une réforme de l'apprentissage et de la formation professionnelle, adossée à un grand plan d'investissement en faveur du développement des compétences et de la formation. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, faisons de la ratification de ces ordonnances une perspective de redressement pour la France. Nous soutenons ce texte qui apportera aux 18 millions de salariés, aux 3 millions d'entreprises et aux 2,6 millions de demandeurs d'emploi que compte

Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le président-rapporteur de la commission des affaires sociales, mes chers collègues, avec l'examen de ce projet de loi de ratification des ordonnances relatives au renforcement du dialogue social, nous arrivons au terme d'un processus qui, à l'origine, avait soulevé pas mal de critiques ou de craintes de la part des partenaires sociaux et du Parlement. Il convient aujourd'hui de reconnaître que cette procédure, annoncée par le candidat devenu Président de la République, s'est déroulée dans des conditions assez satisfaisantes d'échange et de dialogue entre, d'une part, le Gouvernement, et, d'autre part, les partenaires sociaux et les assemblées parlementaires. Si la ligne directrice de ces ordonnances est restée ferme et cohérente, des infléchissements et des améliorations ont pu être introduits tout au long du cheminement de ce texte. J'espère, madame la ministre, que cela pourra encore être le cas lors de la discussion qui s'engage aujourd'hui au Sénat. La plupart des propositions constructives consistent en des amendements de précision ou de simplification, inspirés par la volonté d'élaborer le texte le plus abouti possible. Ces ordonnances s'inscrivent dans le prolongement de la loi du 8 août 2016, dite « loi El Khomri » avec un champ d'intervention plus restreint, mais des dispositions nettement plus réformatrices, notamment en ce qui concerne l'organisation du dialogue social. La démarche globale inclura aussi- il faut mettre ces éléments en perspective -les réformes de l'apprentissage, de la formation professionnelle, de l'assurance chômage et des retraites. C'est à l'issue de ce parcours réformateur qu'il conviendra d'évaluer le nouvel équilibre qui aura été trouvé entre libéralisation et protection, sans doute quelques compléments souhaitables concernant les travailleurs détachés, les nouveaux emplois indépendants ou le renforcement de l'intéressement financier des salariés aux résultats des entreprises.

d'en augmenter le nombre dans les PME et TPE en ouvrant ces accords, en l'absence de délégués syndicaux, aux délégués du personnel et, en dernier ressort, à une consultation directe des salariés, le périmètre à prendre en considération pour évaluer les difficultés d'une entreprise, les contrats de chantier ou d'opération à durée indéterminée, la fusion des instances de représentation des salariés, qui va atténuer l'effet dissuasif de seuil pour les entreprises dont l'effectif atteint 50 salariés,

Cette modification significative du code du travail, en allégeant les contraintes supportées par les entreprises et en réorganisant les outils du dialogue social, stimulera le désir d'entreprendre et d'investir dans notre pays, et favorisera ainsi le développement des entreprises,

Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le président de la commission des affaires sociales, mes chers collègues, six mois, presque jour pour jour, après l'examen du projet de loi d'habilitation, notre assemblée se prononce sur la ratification des cinq ordonnances « pour le renforcement du dialogue social Six mois pour réformer ce qu'on disait irréformable : ce n'est pas un mince succès. Il n'y aura pas de pause dans les réformes d'ampleur dont notre pays a besoin pour retrouver confiance en l'avenir. Le Gouvernement a déjà mis sur le métier de nombreux sujets, notamment celui de la formation et de l'apprentissage, avec la même volonté de concertation et de dialogue.

C'est l'un des rares moments de notre histoire où démocratie sociale et démocratie politique ont marché de concert pour, au final, au travers de ces ordonnances, confier à la société civile un réel pouvoir de fixer des règles du jeu au plus près des réalités des entreprises.

Le 24 juillet dernier, à cette tribune, notre regrettée collègue Nicole Bricq, avec son habituelle acuité, soulignait en ces termes l'enjeu des ordonnances Cette réforme de fond du dialogue social participe d'une bataille culturelle, voire idéologique ; nous savons tous que les batailles de ce genre sont les plus difficiles à mener, parce qu'il faut passer d'une culture conflictuelle à une culture du dialogue. Celui-ci n'exclut pas les confrontations, mais il recherche les points de passage d'accords collectifs. » Pour gagner cette bataille culturelle, il nous faut parier sur l'intelligence collective des entreprises, des syndicats, des salariés et de leurs représentants. C'est pourquoi le coeur de la réforme dont nous sommes saisis donne à la négociation collective, notamment dans l'entreprise, une place sans précédent dans notre histoire sociale. Comme le soulignait Michel Rocard en 2012, « en France, l'essentiel du progrès social doit se faire et s'est toujours fait par la loi. Rien n'est contractuel. » Il ajoutait : « Cela correspond aussi à l'esprit jacobin, qui considère que tout est politique. La société civile disparaît et la société française est obligée d'avancer par coups de sang. Ce qui est très mauvais. Avec le Président de la République, le Gouvernement et la majorité, nous affirmons que notre République sociale est mûre pour accorder une place beaucoup plus importante à la société civile et au droit « négocié Les quatre premiers articles du projet de loi, enrichis par le travail parlementaire, contiennent de grandes avancées pour vivifier le dialogue social. Ainsi, ils établissent une nouvelle architecture conventionnelle d'accorder plus de place à l'accord d'entreprise et de renforcer la branche dans son rôle de définition des conditions de travail, tout en prenant en compte les spécificités des entreprises de moins de 50 salariés. La périodicité et le contenu des consultations et des négociations obligatoires de branche et d'entreprise afin de ménager plus de souplesse et de mieux les adapter aux spécificités du secteur d'activité ou de l'entreprise. La possibilité encadrée d'adopter des accords dans les entreprises de 11 à 50 salariés en l'absence de mandatement La création du comité social et économique, issu de la fusion de trois instances de représentation du personnel, permettra la mise en place d'un dialogue social à la fois plus stratégique, plus concret et moins formel. Ce comité social et économique en conseil d'entreprise doté de la compétence de négociation. C'est une première étape vers ce qui pourrait représenter un modèle de codécision à la française.

Le travail en commission a permis de progresser encore sur de nombreux points. Néanmoins, nous restons en désaccord avec le rapporteur sur certaines dispositions, en particulier la suppression des observatoires départementaux d'analyse et d'appui au dialogue social. Nous présenterons également deux amendements visant à adapter aux réalités du terrain la règle de limitation dans le temps des mandats des élus.

la philosophie de cette réforme, qui n'est pas inspirée par le trompeur selon lequel la complexité et la rigidité du droit du travail seraient les principales responsables de tous nos maux, à commencer par le chômage qui frappe notre pays. ne doit cependant nullement nous empêcher de simplifier, de sécuriser ou d'adapter des mécanismes et des dispositifs qui permettent de pérenniser et de soutenir les entreprises quand la reprise est là.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, comme l'a rappelé Laurence Cohen, le Gouvernement, en procédant par ordonnances et en nous demandant maintenant de ratifier des mesures qui sont déjà appliquées, nous semble mépriser la représentation nationale. Je sais que la majorité sénatoriale s'est ralliée, si ce n'est sur la forme, en tout cas sur le fond à ce projet de loi. Les arguments développés par les uns et les autres n'enlèvent cependant rien à l'opposition frontale du groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste à la philosophie de ce texte. La première ordonnance, qui porte sur la négociation collective, généralise l'inversion de la hiérarchie des normes et donne la primauté à l'accord d'entreprise. Cela pourra conduire à la remise en cause d'avantages acquis, comme le treizième mois ou la prime d'ancienneté. La deuxième ordonnance réduit les prérogatives et les moyens des représentants du personnel. La troisième ordonnance, qui prévoit la barémisation des indemnités prud'homales, ne sécurise que les employeurs et encouragera les licenciements abusifs.

La cinquième ordonnance, sous prétexte de simplification, diminue la protection des salariés soumis à quatre critères de pénibilité, en matière tant de prévention que de réparation.

Ainsi, madame la ministre, vous invoquez l'équilibre de votre texte en vous appuyant sur l'exemple des ruptures conventionnelles collectives. Drôle d'exemple, puisque cette mesure a été introduite par surprise, sans être débattue avec les organisations syndicales ! Drôle de concertation !

ou de son équilibre. Nous n'avons pas la même appréciation : les ruptures conventionnelles collectives chez PSA sont la suite logique des accords de compétitivité, qui se sont tout de même traduits, pour ce groupe automobile, automobile, par la disparition de 25 000 emplois depuis 2013 ! En réalité, vous autorisez des suppressions de postes de travail

de 1 300 embauches en CDI, dont 400 seulement en production, qui réglera les problèmes chroniques de sous-effectif et ceux liés à un intérim durable et sciemment

Lors des auditions menées par la commission des affaires sociales, les organisations patronales n'ont pas caché leur satisfaction

L'arrogance du MEDEF est désormais telle que son représentant s'est même permis d'énoncer devant la commission des affaires sociales des contre-vérités sur la répartition des richesses créées dans l'entreprise, alors que notre pays, de fait, est devenu le plus gros distributeur de dividendes après les États-Unis. C'est cela, malheureusement, qui freine l'investissement productif, et c'est cela qu'il faudrait corriger. En réalité, cette énième réforme du droit

notre groupe votera contre ce texte et proposera des amendements alternatifs visant à s'attaquer aux vrais défis de notre temps : déprécarisation du travail, exercice par les salariés de pouvoirs réels dans la gestion des entreprises, investissement dans l'économie réelle plutôt que financiarisation, responsabilisation des grands groupes envers les PME et TPE, reconnaissance de certaines plateformes numériques comme les véritables employeurs de prestataires prétendument indépendants, exigence de maîtrise du travail et du temps libéré. Pour conclure, nous voterons

Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le président de la commission des affaires sociales, mes chers collègues,

L'épisode malheureux de la loi El Khomri était naturellement dans tous les esprits, qu'il s'agisse du manque de préparation du texte, de l'absence de concertation avec les partenaires sociaux, du recours à l'article 49, alinéa 3, de la Constitution ou encore des très importantes manifestations et autres blocages. Les premières annonces du Gouvernement au sujet de sa réforme du droit du travail ont ravivé ces souvenirs et fait craindre de revivre des semaines de graves perturbations. Le Gouvernement l'a compris, vous l'avez compris, madame la ministre, et vous vous êtes organisée en conséquence. Vous avez d'abord été très claire quant aux ambitions de votre première réforme et sur le fait qu'elle s'intégrait dans un projet cohérent que vous résumiez ainsi libérer l'énergie des entreprises et des actifs, tout en donnant de nouveaux moyens concrets à chacun de trouver sa place sur le marché du travail et de construire son parcours professionnel. Les ordonnances pour le renforcement du dialogue social sont la première étape de la mise en oeuvre d'un plan qui se poursuivra, au printemps prochain, par la réforme de l'assurance chômage, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Le droit du travail est donc assoupli, simplifié, sa définition ramenée au sein des entreprises, échelon le plus pertinent. En parallèle, la protection des salariés est renforcée afin qu'eux aussi puissent s'adapter aux transitions professionnelles liées à une économie en constante mutation. qui sera atteint grâce à la modernisation de l'offre de formation professionnelle et de l'apprentissage, mais également par le biais de la réforme de l'assurance chômage. Vous avez ensuite mis en oeuvre une méthode : celle du dialogue et de la concertation.

Le recours aux ordonnances n'est pas du goût des parlementaires que nous sommes, vous l'avez bien compris, mais vous avez fait le choix de la réactivité pour relancer notre économie ; nous respectons ce choix. Nous avions passé des semaines à discuter de la loi El Khomri, et nous avons validé les contours des ordonnances que vous nous demandez maintenant Vous vous êtes saisie d'un outil que vos principaux détracteurs n'ont jamais hésité à utiliser, et vous avez envoyé rapidement un premier signal fort. Vos prochaines réformes suivront la procédure classique, et nous aurons de très nombreuses heures de séance publique pour nous exprimer et exercer pleinement notre droit d'amendement. J'en viens plus précisément au projet de loi de ratification que nous examinons aujourd'hui. Parmi les principales mesures que je tiens à mettre en exergue figure la réorganisation de l'architecture conventionnelle au profit des accords d'entreprise. Vous permettez enfin aux entreprises d'adapter les règles à leur activité. Les branches ne sont pas pour autant oubliées, bien au contraire, puisque leur rôle est clarifié et conforté. Elles pourront prendre en compte les besoins spécifiques des petites et moyennes entreprises.

La définition des règles à l'échelon de l'entreprise se fera dans le cadre d'un dialogue social rénové, donnant plus de place à la consultation des salariés. Les possibilités sont nombreuses, en fonction de la taille de l'entreprise et de la présence ou non de représentants élus du personnel ou de délégués syndicaux. L'objectif est clair : encourager le dialogue et la définition concertée des règles de travail. Je salue également la création du comité social et économique, issu de la fusion des délégués du personnel, du CHSCT et du comité d'entreprise. Les prérogatives de chacune de ces institutions ne seront pas réduites ; il s'agit au contraire de les renforcer grâce à une plus forte visibilité. Les entreprises n'auront plus la crainte de franchir le seuil fatidique des 50 salariés. L'ordonnance relative à la prévisibilité et à la sécurisation des relations du travail comporte sans doute les mesures les plus controversées de cette réforme : le plafonnement des indemnités prud'homales et la rupture conventionnelle collective. Le plafonnement des indemnités prud'homales avait cristallisé les oppositions à la loi El Khomri, conduisant le gouvernement d'alors à renoncer et à ne proposer qu'un barème indicatif. Votre réforme, madame la ministre, va jusqu'au bout de la logique, tout en prévoyant les verrous nécessaires. Elle offrira à la fois de la visibilité pour les employeurs et la garantie d'une justice protectrice pour les salariés. La rupture conventionnelle collective, particulièrement médiatisée et caricaturée ces derniers temps, offre également de la souplesse aux entreprises dans la gestion de leur masse salariale et évitera les licenciements massifs issus d'un défaut d'anticipation.

qui en est le bras armé, est toujours abordée de manière parcellaire, sans vision d'ensemble. Non seulement cette filière subit une importante perte perte d'attractivité, mais son intérêt n'est pas non plus compris, voire admis, par les entreprises, qui, rappelons-le, la financent. La médecine du travail doit pourtant être vue comme une contrainte pour les entreprises, mais bien comme une alliée de la productivité de leurs salariés. En outre, elle s'intègre parfaitement dans la responsabilité sociale des entreprises. Madame la ministre, le groupe Union Centriste soutient ce qui n'est qu'une première étape de votre réforme de notre modèle social. Nous demeurerons néanmoins attentifs et surtout particulièrement exigeants quant à la mise en oeuvre des mesures de protection et d'accompagnement des salariés. de vous remercier

Nous allons débattre et tenter d'apporter des améliorations à un texte qui, selon l'essayiste Mathieu Laine, grand zélateur du Président de la République, « va plus loin que les réformes de Chirac, Sarkozy et Hollande réunies » : c'est édifiant, non ?

cependant plus qu'un fossé qui sépare le verbe de la réalité. Il y a un océan entre la suppression de la taxe d'habitation et sa compensation encore indéfinie, entre le discours et la vérité sur le pouvoir d'achat ou sur sur la résorption, plus qu'improbable, du déficit budgétaire, que les charges reportées sur 2019 vont considérablement creuser. La réforme du code du travail relève parfaitement de ce hiatus entre les déclarations lénifiantes et les effets toxiques des ordonnances. Ainsi, avant même qu'aient été mesurés les effets de la loi El Khomri, vous en bouleversez l'économie. Les syndicats, unanimes, condamnent la régression représentée par un texte mis en place avant toute évaluation du précédent. Ne condamniez-vous pas vous-même les cadres législatifs ou fiscaux trop changeants ? Vérité quand cela vous arrange, erreur sinon ... Nous aurions pu vous rejoindre sur la double ambition déclarée : favoriser la compétitivité des entreprises et sécuriser l'emploi. Hélas, si le premier volet est largement satisfait- les organisations patronales vous disent merci -, c'est au détriment du second. De tristes illustrations viennent douloureusement confirmer nos inquiétudes. Ainsi, Castorama, réclamait des licenciements plus souples et le plafonnement des indemnités prud'homales, et devait en retour créer 5 000 emplois. Le groupe a obtenu ce qu'il attendait, et déménage son siège en Pologne PSA fait de larges bénéfices- nous nous en réjouissons -et profite du dispositif de rupture conventionnelle collective pour se séparer de 1 300 salariés, parmi les plus âgés, et les remplacer par autant de jeunes aux salaires moins élevés. moins élevés. Comme lui-même le titrait sans nuances, « Le Gouvernement n'écoute que le MEDEF ». En réalité, ces ordonnances font du licenciement un mode banal de gestion, précarisent les salariés, durcissent les conditions de travail et sacrifient la santé et la sécurité des personnels. Ainsi, les accords d'entreprise pourront, en dehors de l'intervention de toute représentation syndicale, décider de modifier les conditions et les horaires de travail, y compris de nuit, la rémunération, par la modulation ou la suppression des primes, les abondements pour heures supplémentaires.

de désaccord d'un salarié dont on aura ainsi modifié le contrat de travail, celui-ci pourra être licencié sans que le caractère « réel et sérieux » du motif puisse être contesté. Hier, le rachat d'une entreprise imposait au repreneur de reprendre l'ensemble du personnel. Dorénavant, le vendeur pourra spéculer sur le prix en engageant, avant cession, les procédures de licenciement.

que l'exigent les nécessités de fonctionnement de l'entreprise ». On ne saurait faire plus flou ni plus large ! Toute tentation d'exiger des sacrifices supplémentaires pourra se donner

bien entendu, puisqu'il faut faire du licenciement une opération banale et sans risque pour l'employeur, les délais de recours contre une décision jugée injuste ou arbitraire sont raccourcis. la ministre, vouloir intensifier le dialogue social, mais un dialogue ne peut exister qu'entre deux interlocuteurs égaux en droit. Aussi votre déclaration relève-t-elle plus de l'incantation que de la réalité. Désormais, dans la majorité des entreprises de moins de 50 salariés, de moins de 50 salariés, la participation syndicale ne sera plus assurée. La relation de subordination, donc la menace, réelle ou supposée, qui pèsera sur les épaules des salariés élevés au rang de négociateurs, conduira forcément à une négociation pipée, ce ce qui ne servira ni l'entreprise ni les travailleurs qui en font le dynamisme. Quant au référendum à la main du patron, il fait l'unanimité contre lui. On ne peut imaginer un seul instant une négociation équilibrée quand les questions posées n'auront fait l'objet d'aucune discussion préalable, tandis que la réponse, réduite à « oui » ou à « non », exclut », exclut toute adaptation. Le périmètre même d'un tel référendum ne va pas sans poser question quand tous les salariés ne sont pas concernés ou victimes potentielles.

Contrairement aux promesses faites, l'obligation d'instaurer une commission spécifique n'existera qu'à partir de 300 salariés. En outre, cette commission perdra ce qui faisait l'efficacité du CHSCT, à savoir la personnalité juridique et la possibilité d'ester en justice. Voilà la sécurité et la santé ramenées au rang de préoccupations subalternes les salariés seront précarisés. Il faut être poète pour qualifier de CDI des contrats de chantier. La possibilité de généralisation de ces contrats par les branches risque d'augmenter le nombre de travailleurs précaires,

aux fondements de notre droit, qui, jusqu'à présent, exigeaient que chacun puisse bénéficier d'une juste et complète réparation, obligatoirement individualisée. Le juge

Villepin, ce contrat première embauche que nous avions tant combattu. Eh oui ! Nous aurons l'occasion de le montrer. Circonstance « exténuante », acharnement supplémentaire, le juge peut dispenser de l'application de l'effet rétroactif à compter de la date du licenciement et intégrer des indemnités légales dans la réparation du préjudice. Les ordonnances ne se bornent pas à supprimer une grande partie des moyens d'alerte sur les risques pour la santé et la sécurité par la suppression des CHSCT, elles s'en prennent à la prévention et à la réparation des handicaps et maladies liés

ordonnance-Arlésienne pourrait apparaître brusquement et dessaisir le Parlement de ses prérogatives. Sans doute n'est-ce là qu'une rumeur ! Il va de soi que le Gouvernement ne saurait agir de la sorte ... Madame la ministre,

Aujourd'hui, fait rare dans notre histoire, c'est une régression grave que vous nous proposez d'approuver. Nous voterons donc contre votre projet

Monsieur le président, madame le ministre, monsieur le président de la commission, mes chers collègues, le président de notre groupe, Claude Malhuret, s'est déjà exprimé sur l'opportunité de ce projet de loi et l'importance de ces ordonnances. Je n'y reviendrai donc pas. Il me paraît important de souligner que cette réforme, pourtant difficile, a été menée dans un climat serein,

simplifient certaines règles qui constituaient indéniablement un frein au développement de l'emploi, apportent de la flexibilité et, ainsi, adaptent notre législation du travail à l'évolution de notre économie sans précariser les salariés. Les règles relatives à la négociation collective sont clarifiées grâce à une articulation cohérente entre accords de branche et accords d'entreprise, une place importante étant donnée

par 50 % des syndicats. Monsieur le président, madame le ministre, mes chers collègues, le groupe Les Indépendants-République et Territoires est favorable à ces ordonnances. En France, l'emploi industriel a reculé de 25 % en quinze ans. Notre législation, qui se voulait vertueuse en étant très protectrice envers les salariés, pouvait, par excès de contraintes, freiner le développement de l'emploi. Dans ce contexte, il fallait faire évoluer les règles qui régissent notre économie pour aller vers le plein-emploi, sans précariser les salariés, mais en visant une augmentation du nombre d'embauches en CDI dans les entreprises. Après l'adoption de ces ordonnances et la baisse des charges,

La parole est à Mme Catherine Deroche, pour le groupe Les Républicains. Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, nous arrivons à la dernière étape du processus d'adoption des ordonnances. J'espère qu'un accord pourra être trouvé sur les dispositions proposées en commission par le rapporteur.

sur les projets de loi dits « Rebsamen », « Macron » ou « El Khomri » ou de textes tels que la proposition de loi relative aux entreprises de notre collègue Alain Chatillon. Je rappellerai nos positions, pour apporter des précisions sur ce que nous soutenons et sur ce que nous ne soutenons pas. En effet, si nous souscrivons au projet global, le Gouvernement est loin d'avoir supprimé tous les freins au développement de nos entreprises, alors que le Président de la République présente ces ordonnances la principale réforme de son quinquennat. Tout d'abord, en matière de dialogue social, nous souhaitions la primauté des accords d'entreprise, parce qu'il est important que les décisions soient prises au plus près du terrain, d'un commun accord entre les acteurs concernés.

Étendre la primauté des accords de branche est judicieux dans certains domaines, mais, dans d'autres, cela restreindra le champ des possibles pour les entreprises. Ce sera notamment le cas pour les contrats de mission, dont le Gouvernement affirme pourtant vouloir favoriser le développement. D'autres dispositions concernant les accords de branche sont au contraire judicieuses, comme l'obligation de prévoir des dispositions spécifiques qui tiennent compte de la réalité des TPE-PME. Concernant précisément les TPE-PME, nous nous réjouissons que soit favorisé un dialogue social direct, avec la possibilité, pour les entreprises de moins de 50 salariés, de négocier avec un élu du personnel en l'absence de délégué syndical, et, pour les TPE de moins de 20 salariés, de consulter le personnel en l'absence de représentant élu. De même, notre groupe demandait depuis des années une simplification des instances représentatives du personnel. Celle-ci est réalisée aujourd'hui par la fusion des trois instances d'information au sein d'un comité social et économique. Plusieurs mesures avaient été également proposées par notre groupe concernant la sécurisation des relations de travail. Je pense d'abord au plafonnement des indemnités en cas d'absence de cause réelle et sérieuse d'un licenciement

Je précise que, sur ces deux sujets, les ordonnances ne font qu'appliquer des règles qui sont suivies par la majorité des autres pays européens. Je citerai également l'harmonisation des accords dits « offensifs » et « défensifs », qui permettent aux entreprises d'anticiper et de s'adapter rapidement aux évolutions à la hausse ou à la baisse du marché, ou encore la création de conventions collectives reprenant le principe des conventions individuelles créées par notre majorité que les entreprises et leurs salariés s'étaient rapidement appropriées. Enfin, le dossier de la pénibilité trouve une issue, même si le sujet est loin d'être clos. Pour ma part, je crains les effets du transfert du financement à la Caisse Malgré toutes ces dispositions favorables au développement de l'activité, à l'issue de ces quelques mois de préparation des ordonnances, les retours du terrain dans nos circonscriptions montrent que les entreprises ne sont toutes convaincues par l'action du Gouvernement. J'y vois plusieurs explications. Si des incertitudes sont levées, un sentiment de fragilité face aux nombreuses contraintes administratives et fiscales auxquelles les entreprises sont soumises aujourd'hui L'action du Gouvernement comporte des contradictions. Par exemple, si des dispositions ont été prises pour que les entreprises puissent anticiper le coût d'un licenciement, les indemnités légales de licenciement ont parallèlement été augmentées de 25 Le décret d'application a d'ailleurs été pris quelques jours seulement après la publication des ordonnances. Cela n'est pas de nature à rétablir la confiance, d'autant que l'essentiel manque. Comme vient de le souligner le président Retailleau, le Gouvernement n'a pas souhaité inclure dans les ordonnances la réforme pourtant capitale des seuils sociaux et fiscaux, ni évoquer la question du temps et du coût du travail. Notre vote positif s'accompagnera donc de nombreuses réserves et traduit une position d'attente. Les Français ont voté aux élections présidentielles pour une rupture, pour une véritable politique de développement de l'activité et de l'emploi, avec les réformes structurelles et les choix budgétaires que cela implique. Même si ce texte va dans le bon sens, je ne perçois pas, pour le moment, le courage politique que nécessitent de tels changements. Je le regrette sincèrement. La discussion

Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le président de la commission des affaires sociales, mes chers collègues, la publication et l'entrée en vigueur progressive des cinq ordonnances confirment les ambitions libérales du Gouvernement en matière d'emploi et de dialogue social. Ces ordonnances relèvent d'une logique d'abord comptable qui, plutôt que de favoriser l'emploi, renforce les moyens de le réduire, privilégie la flexibilité plutôt que la justice sociale. Le rejet exprimé par l'ensemble des syndicats de salariés est, en lui-même, assez éloquent quant à l'esprit de ces textes qui ont fait l'objet d'une concertation menée au pas de course et qui, de plus, ne sont accompagnés d'aucune étude d'impact. Ces ordonnances pourraient être qualifiées, selon l'expression forgée par le célèbre juriste universitaire Alain Supiot, de nouveau « produit législatif » proposé sur le marché international des normes. Il porte de sérieux reniements de notre modèle social et économique. La loi semble détournée de son objectif premier, à savoir la fixation des conditions de justice entre le salarié et l'employeur.

Des réponses novatrices furent élaborées pour adapter notre droit à la numérisation du travail. Je pense au compte personnel d'activité, au droit à la déconnexion, à la prise en compte de la pénibilité, aux congés spéciaux, aux emplois saisonniers, etc.

Rappelons que ce nouvel outil permet aux entreprises de licencier sans justification économique et à moindres frais, en évitant les contraintes d'un plan de sauvegarde pour l'emploi, dispositif qui limitait jusqu'à présent le nombre des licenciements. les salariés, la RCC les prive de leur droit au contrat de sécurisation, qui leur offrait un meilleur suivi post-licenciement et leur assurait pendant un an une indemnité plus élevée que l'indemnité de base. La conjoncture favorable pour l'emploi que nous connaissons depuis quelques mois et dont il semble difficile de ne pas attribuer la paternité au précédent quinquennat la paternité suffira-t-elle à masquer les aspects délétères de cette mesure pour les parcours professionnels de nos concitoyens ? Maintes dispositions, évoquées par mes collègues, constituent autant de renoncements et d'innovations régressives, qui tendent à une généralisation de la précarité et à un affaiblissement du dialogue social. autres mesures, la barémisation impérative des indemnités prud'homales, qui remet en question le principe fondamental de « réparation intégrale » des préjudices subis, la limitation du périmètre d'appréciation du motif économique, qui permettra aux multinationales implantées sur notre territoire de procéder plus facilement à des licenciements massifs, l'assouplissement des obligations de reclassement dans le cadre d'un licenciement économique, le contournement des syndicats par l'employeur dans les petites entreprises de moins de 20 salariés l'instauration d'un référendum à la main du patron, la suppression du CHSCT, créé par les lois Auroux de 1982, l'intégration de cette instance sanitaire dans le comité social et économique la dépossédant, en vérité, de sa capacité à ester en justice et à recourir à des expertises. Toutes ces mesures ne traduisent-elles pas la volonté du Gouvernement de parier sur la dérégulation au détriment des protections salariales, uniquement perçues comme des contraintes ? Où est l'humain dans tout cela ? L'esprit de ces ordonnances est trop éloigné de la réalité humaine et psychologique des salariés. La création des « CDI de chantier ou d'opération » n'est-elle pas une innovation juridique visant à précariser encore un peu plus le monde du travail, déjà marqué par l'importance du recours aux CDD et à l'intérim ? autre point auquel je demeure très attentive : la prévention de la pénibilité. Le dispositif a été souvent qualifié d'« usine à gaz », et les syndicats étaient eux-mêmes conscients de la perfectibilité des référentiels. au lieu de tendre vers un système coconstruit avec l'ensemble des partenaires sociaux, le Gouvernement a manifestement cédé aux arguments des organisations patronales. Le retrait de quatre facteurs de risque liés à des contraintes physiques marquées,

Par ailleurs, le nouveau système entré en vigueur au 1 octobre dernier prévoit qu'il faudra avoir été atteint par une pathologie avant la date de départ à la retraite. Ne s'agit-il donc pas là d'un renversement de la logique même de prévention des risques ? des risques ? Jusqu'alors, le salarié acquérait des droits « à raison de son exposition sans exigence d'une affection » ou d'un taux minimal d'incapacité permanente partielle. Alors qu'a été déposée une proposition de loi portant création d'un fonds d'indemnisation des victimes des pesticides, les fiches d'exposition aux risques chimiques, notamment à l'amiante, instaurées sous Lionel Jospin sont purement et simplement supprimées. Nous ne pouvons être partisans d'une simplification du droit allant à l'encontre de la santé des salariés.

Pour nous, l'entreprise n'est pas seulement la propriété de l'employeur, ni uniquement le lieu de la production de biens et de services ; c'est aussi un lieu de création collective et d'interaction sociale où l'être humain doit pouvoir se réaliser et se révéler. Le dialogue social est un élément essentiel du nécessaire rééquilibrage des rapports de force existants au sein de cette organisation humaine., la philosophie défendue ici par le Gouvernement relève d'une idéologie verticale de l'entrepreneuriat envisageant les règles comme des contraintes et les droits comme des coûts. À l'heure de la révolution numérique, il est regrettable de voir réapparaître en France une vision passéiste du dialogue social, selon laquelle le bien-être des salariés serait contre-productif et altérerait la performance économique. L'humain n'est pas une simple variable d'ajustement. Au regard de cet écueil idéologique, il est également fort regrettable de ne relever aucune mesure d'anticipation des grandes mutations du travail : ubérisation, recrudescence des mini-jobs, multiplication des contrats excessivement précaires. Les salariés étaient pourtant dans l'attente d'une meilleure sécurisation des parcours professionnels. Madame la ministre, en raison de l'adoption d'une sixième ordonnance présentée en conseil des ministres le jour de l'examen du rapport de la commission des affaires sociales du Sénat, soit le 20 décembre dernier, et dans l'attente de la publication de la septième, toujours en préparation, nous considérons que les conditions ne sont pas réunies pour travailler correctement et avoir un débat approfondi permettant de mesurer les tenants et les aboutissants de l'ensemble des dispositions proposées par le Gouvernement. Bien que décrite comme une « ordonnance balai », ce qui sous-entend que ce texte n'apporterait que des précisions d'ordre technique, il s'avère que la sixième ordonnance, qui, faut-il le préciser, n'a fait l'objet d'aucune concertation, pose de nombreuses questions qui ne pourront pas être débattues dans de bonnes conditions.

Je pense notamment aux nouvelles prérogatives octroyées au « conseil d'entreprise », qui serait seul compétent pour négocier tout type d'accord d'entreprise, privant ainsi les délégués syndicaux du pouvoir de négocier.

parlementaire ne saurait éluder cette question. Certaines obligations d'information des salariés licenciés sont également purement et simplement supprimées. Il conviendrait pourtant d'en débattre et de donner au Parlement le temps nécessaire à l'examen de ces ordonnances tardives ; la septième n'est d'ailleurs même pas encore connue. La procédure par ordonnances est une pratique dérogatoire permise par l'article 38 de la Constitution. Nous en convenons, mais avec une certaine amertume.

Pouvez-vous nous dire, madame la ministre, au regard de l'avancement du travail législatif en cours, quand le Parlement disposera de l'ensemble des éléments pour jouer son rôle constitutionnel de législateur ?

je voudrais, en préambule, féliciter M. Patrick Kanner, élu ce matin président du groupe socialiste et républicain.

Monsieur le Premier ministre, vous avez annoncé la semaine dernière votre décision d'abandonner le projet de construction de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes.

Désormais va s'ouvrir la phase de l'évacuation de la ZAD, qui regroupe, je le rappelle, des occupants sans droit ni titre. Vous avez choisi une double approche, en fixant au printemps prochain le dernier délai d'évacuation des lieux tout en exigeant le déblocage immédiat des routes. Pour notre groupe, il n'est pas acceptable que des expressions minoritaires bloquent tout projet, au mépris des processus démocratiques. C'est pourquoi nous attendons des précisions sur le calendrier que vous mettrez en oeuvre. Mais une question plus large se pose : celle de l'intangibilité de l'ordre républicain dans les autres ZAD placées sous la

quelles mesures comptez-vous prendre pour assurer le maintien de l'ordre républicain et faire respecter l'autorité de l'État en mettant fin à l'existence de ces zones de non-droit ?

Il se trouve que, au cours de la législature précédente, les conditions dans lesquelles certains occupants peuvent être considérés comme résidents

C'est, au fond, un art d'exécution : nous devons faire en sorte de réagir suffisamment tôt pour que jamais nous ne nous trouvions de nouveau dans une situation où la division soit telle que le projet ne puisse plus avancer. C'est une tâche difficile qui est

Les hauts fonctionnaires se sont constitués en caste. [ ...] Il n'est pas acceptable qu'ils continuent à jouir de protections hors du temps. » Ainsi parlait le révolutionnaire Emmanuel Macron lors de sa campagne élyséenne.

Ma question est simple : quand le Gouvernement envisage-t-il de mettre fin à cette situation, en commençant par publier les montants des salaires des quelque 600 hauts fonctionnaires recevant annuellement plus de 150 000 euros nets, soit le montant de l'indemnité du Président de la République ?

ce qui relativise le procès fait actuellement à la fonction publique. Il faut aussi souligner que le niveau des responsabilités confiées et les qualifications requises justifient, dans l'immense majorité des cas, les traitements versés. Le déploiement du régime indemnitaire, qui tient compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel, permet progressivement de franchir une nouvelle étape dans la transparence et la cohérence des rémunérations. Les sous-directeurs et chefs de service des administrations centrales sont régis par ce dispositif depuis le début de 2017, et les emplois de direction de l'administration territoriale de l'État depuis le mois de juillet de la même année. Ainsi, le plafond de leur rémunération indemnitaire est fixé à 74 000 euros.

Ce travail est engagé depuis le début des années 2000. Aujourd'hui, ne subsistent que sept situations relevant d'un droit que l'on peut qualifier d'exorbitant ; elles sont en cours de règlement. Le Gouvernement a prévu l'extinction de ces dispositifs au 1 janvier 2019, plutôt qu'en 2023, comme précédemment programmé.

Monsieur le secrétaire d'État, si je comprends bien, la réponse à ma question, c'est : « Touche pas à ma bureaucratie céleste, touche pas au grisbi ! En fait de révolution annoncée, ce n'est même pas une émeute, c'est un simple produit marketing, lancé pour se faire mousser

Cette situation est aussi dramatique qu'inquiétante, et ce à plus d'un titre. Elle est dramatique, parce que cette zone gérée par les Kurdes était l'une des rares parties du pays à avoir été épargnée jusqu'alors par les combats. l'est également parce que ce conflit, complexe du fait du nombre et de l'opacité des acteurs en présence, charrie depuis ses origines les germes d'un embrasement régional. En intervenant, troupes au sol à l'appui, Ankara prolonge le conflit et bouscule le rapport de force au sein des forces libres syriennes, éloignant un peu plus les perspectives de paix. Le président Erdogan, reçu par l'Élysée en début d'année, a d'ailleurs déclaré qu'« il n'y aura pas de retour en arrière Pourtant, mes chers collègues, l'YPG est connue pour ses faits d'armes contre l'État islamique et a contribué largement à la défaite de ce dernier sur le terrain. C'est donc une composante essentielle du front commun contre le terrorisme qui est aujourd'hui attaquée. inquiétante, enfin, parce qu'il s'agit d'une intervention militaire d'un État membre de l'Alliance atlantique menée en violation des règles les plus élémentaires du droit international. La France a été à l'initiative de la tenue d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations unies sur le sujet.

soit stoppée et qu'un cessez-le-feu intervienne dans les plus brefs délais, alors que les États-Unis semblent se désengager totalement de cette région. Il y a urgence, monsieur le Premier ministre.

la défaite attendue de Daech risque de se traduire par une mutation des conflits : Turcs contre Kurdes, Kurdes contre Arabes,

L'opération turque intervient à un moment où la situation humanitaire dans la région, du fait de la guerre terrible qui s'y déroule depuis maintenant de longues années, est incroyablement fragile. Le régime et ses alliés conduisent des bombardements indiscriminés contre les populations à Idlib, 400 000 civils sont assiégés dans l'enclave de la Ghouta, près de Damas. À notre demande, le Conseil de sécurité s'est saisi hier de cette situation. Nous avons appelé la Turquie à la retenue.

Cela consiste à inciter les automobilistes qui circulent sur les grands axes aux heures de pointe à utiliser d'autres modes de déplacement ou à reporter leurs trajets en dehors de ces périodes. Une incitation financière de 2 euros par trajet évité leur sera ainsi proposée. Cette initiative, appelée « écobonus-mobilité », est le projet phare du pacte État-métropole signé le 17 février 2017. Il s'agit d'une réelle occasion d'innover pour trouver des solutions concrètes et rapides aux phénomènes de congestion routière constatés dans toutes les grandes agglomérations françaises.

Pour donner aux collectivités les moyens de construire une mobilité durable et de rendre les villes de nouveau respirables, la loi autorise depuis 2010 l'expérimentation des péages urbains, pour l'expérimentation des péages urbains, pour trois ans. Le principe de ce dispositif est simple : permettre aux collectivités qui le souhaitent d'inventer des solutions incitant au report modal, à l'usage des transports en commun ou du vélo.

un bonus aux conducteurs qui acceptent de recourir à d'autres modes de transport que la voiture pendant les heures de pointe. D'autres mesures, visant notamment à simplifier la création de voies dédiées aux covoitureurs sur les axes d'entrée dans les grandes agglomérations,

Est-ce là, monsieur le Premier ministre, votre conception de l'aménagement du territoire ? Vous avez pris une décision, il vous faut désormais prendre vos responsabilités : que ferez-vous pour accompagner le désenclavement de l'Ouest et des Pays de la Loire ?

Oui, mercredi dernier, j'ai pris une décision. Ce n'était pas facile. Elle s'est fondée sur l'ensemble des éléments en ma possession au moment où j'ai dû la prendre

mise en place d'une meilleure connexion aux grandes infrastructures aéroportuaires et aux flux de développement économique. La question est posée.

Il faudra voir dans quelle mesure les propriétaires des infrastructures existantes à Rennes, à Nantes, à Lorient et, de façon générale, dans le Grand Ouest pourront mettre en réseau leurs équipements et les développer.

et les opérateurs nous permettra de dessiner des solutions d'investissement pour améliorer la desserte aérienne. S'agissant de la desserte ferroviaire, il faudra voir dans quelles conditions il est possible de rejoindre les grandes plateformes aéroportuaires.

Union Centriste. Le Président de la République a manifesté hier, à l'occasion de son déplacement chez Toyota et de sa rencontre à Versailles avec 140 patrons de grandes entreprises, sa volonté de défendre l'attractivité de la France et de soutenir l'industrie française. Il va de soi que le patrimoine industriel historique présent sur notre territoire doit bénéficier du même soutien. C'est pourquoi, madame la secrétaire d'État, je me permets de vous interroger sur l'avenir du groupe Vallourec. En 2016, le Gouvernement avait participé à une recapitalisation de ce groupe à hauteur de plus de 500 millions d'euros, par l'intermédiaire de la Banque publique d'investissement, la BPI, en contrepartie de l'engagement pris auprès de M. Macron, alors ministre de l'économie, de ne fermer aucun site de production. Cet engagement n'était que verbal. On me dit que c'est normal. Habituée que je suis au formalisme entourant le versement des subventions aux collectivités, j'ai beaucoup de mal à l'admettre

À Cosne-sur-Loire, dans la Nièvre, département dont je suis élue, le site de fabrication de tubes sans soudure n'est pas repris par le groupe américain NOV et 120 emplois sont menacés à très court terme. Dans le Nord, sur le site historique de Valenciennes, où Vallourec est partenaire d'Ascométal, la reprise n'attend plus, pour être finalisée, qu'un engagement officiel de l'État. Derrière Vallourec, ce sont des bassins d'emploi et des sous-traitants qui pourraient être fragilisés, à Montbard par exemple. Certains dossiers présentent un caractère d'urgence absolue. L'État est désormais l'actionnaire principal de Vallourec. Il a consenti en 2016 d'énormes efforts financiers. Madame la secrétaire d'État, pouvez-vous nous confirmer la volonté forte, concrète et immédiate de l'État, d'une part, de soutenir ce fleuron national qu'est l'aciérie française, d'autre part, d'exiger du groupe Vallourec qu'il respecte les engagements pris voilà quelques mois ? La parole

en effet un acteur industriel important sur notre territoire, employant 4 000 salariés en France. Comme vous le savez, cette entreprise a été frappée de plein fouet

par cette décision. Vallourec a annoncé son intention de les mettre en vente et approche actuellement plusieurs partenaires potentiels. Je vous confirme que le Gouvernement est attaché

Le suivi de ce dossier a été confié à Jean-Pierre Floris, délégué interministériel aux restructurations d'entreprises. Il recevra demain les élus du territoire de la Nièvre et se rendra à Tarbes en cette fin de semaine. La parole

et des postes, l'ARCEP, annonçait la signature d'un accord historique visant à généraliser « une couverture mobile de qualité pour l'ensemble des Français ». L'ensemble des Français ? Non, pas exactement, puisque cet accord ne concerne en réalité que la France hexagonale et la Corse Les outre-mer, comme souvent, ont été écartés, car les opérateurs y seraient différents, auraient des fréquences différentes et seraient soumis à des obligations distinctes par territoire. Monsieur le ministre, si je peux entendre ces raisons, les mots n'en ont pas moins un sens, et lorsque l'ARCEP se prévaut d'un accord historique pour tous les Français, nos concitoyens ultramarins sont en droit de s'interroger. À vrai dire, il leur suffit de consulter le site pour comprendre pour comprendre qu'ils ne sont visiblement pas des Français comme les autres, la carte de la France se limitant, là encore, à l'Hexagone et à la Corse. Les besoins sont pourtant bien réels. Si c'est bien de la Guyane que nos satellites de communication sont lancés, le coût des forfaits y reste très élevé et la couverture en téléphonie mobile extrêmement défaillante, en particulier dans les communes isolées et sur les routes nationales. Certes, des efforts sont faits. L'attribution en 2016 de nouvelles fréquences aux opérateurs ultramarins a permis de commercialiser des services mobiles à très haut débit. Mais, là encore, les engagements des opérateurs seront-ils à la hauteur ? Rappelons que, en 2015, l'ARCEP avait dû retirer leurs fréquences à trois d'entre eux suite à des retards de déploiement et de paiements. Dans ce contexte, nous ne pouvons que déplorer, voire dénoncer, le fait que nos territoires ne soient pas, avec leurs particularités de marchés respectives, inclus pleinement dans le champ d'un accord aussi ambitieux. Monsieur le ministre, vous le savez, le défi de la résorption de la fracture numérique que nous avons à relever ensemble est immense, mais aussi fondamental. C'est pourquoi je souhaiterais avoir des précisions sur la stratégie que le Gouvernement entend déployer outre-mer pour renforcer les obligations des opérateurs et mettre fin, une bonne fois pour toutes, aux zones blanches. La parole

pour soutenir la couverture en internet fixe des huit territoires ultramarins. Pour la Guyane, une enveloppe supplémentaire de 40 millions d'euros va être mobilisée. Ensuite, en matière de téléphonie mobile, effectivement, les opérateurs ne sont pas identiques. Ils utilisent des fréquences différentes, avec des calendriers adaptés, et sont soumis à des obligations distinctes par territoire. Un travail est en cours avec l'ARCEP pour identifier les besoins spécifiques, déployer des outils adaptés et arriver à une couverture de qualité généralisée selon le même calendrier que pour le territoire hexagonal. Je tiens à l'affirmer Nous réunirons prochainement les collectivités et les opérateurs concernés pour préciser la feuille de route et voir comment les futures attributions de fréquences outre-mer peuvent constituer un outil pertinent pour renforcer les obligations des opérateurs mobiles. Ce chantier sera inscrit dans les Assises des outre-mer.

turque dans la province kurde syrienne d'Afrin, conduite en violation du droit international. Alors que la coalition internationale affronte, dans la province d'Idlib, l'ex-Front al-Nosra, la branche syrienne d'Al-Qaïda, les forces turques bombardent l'enclave kurde d'Afrin, située au nord de la ville martyre d'Alep. Depuis dimanche, une intervention terrestre est en cours et les correspondances font état de nombreuses victimes civiles. La Turquie mène l'assaut contre l'une des rares villes syriennes qui a, jusqu'ici, échappé à la destruction et servi de refuge à des milliers de déplacés syriens, une ville dont le seul crime est d'être dirigée par des forces kurdes. par des forces kurdes. Or ces forces sont nos alliées dans la guerre contre Daech. Ce sont elles qui, à Kobané, ont infligé une défaite sans appel à Daech. Elles ont mis hors d'état de nuire des milliers de djihadistes et participé à la libération de tous les territoires syriens occupés par Daech, y compris Rakka, capitale du prétendu califat. Alors que l'engagement des Kurdes à nos côtés n'est plus à démontrer, nous savons aussi que des parlementaires et des maires kurdes, élus démocratiquement, sont aujourd'hui emprisonnés en Turquie. Monsieur le Premier vous avez à raison saisi le Conseil de sécurité de l'ONU, qui s'est réuni à huis clos mais dont aucune mesure ne semble être sortie. Nous connaissons votre attachement à soutenir ceux qui combattent pour la liberté. Pouvez-vous nous dire, monsieur le Premier ministre, quelle est la position de la France à l'égard de nos alliés kurdes ? Allons-nous demander le retrait de l'armée turque et l'arrêt immédiat de l'intervention à Afrin ? Peut-on considérer qu'appeler la Turquie à la retenue après une réunion du Conseil de sécurité soit suffisant au regard de la gravité de la situation sur place ?

Vous avez évoqué les civils aujourd'hui menacés : ce sont 400 000 femmes, hommes, enfants qui sont assiégés dans l'enclave de la Ghouta, près de Damas. Vous l'avez dit, à la demande de la France, le Conseil de sécurité s'est saisi hier de cette situation humanitaire.

Ces détenus savent faire preuve de ruse et de dissimulation pour tromper les surveillants et les personnels pénitentiaires d'insertion et de probation. Dans un passé récent, des programmes spécifiques ont été mis en place, tel le regroupement de ces détenus au sein de quartiers. Au vu de ses résultats infructueux, cette politique a été abandonnée à l'automne 2016. unies vient de tirer la sonnette d'alarme en adressant une série de recommandations eu égard aux atteintes aux droits de l'homme commises dans l'Hexagone. Elle a appelé la France à améliorer la gestion de ses prisons dans un contexte de surpopulation carcérale.

? Enfin, pouvez-vous nous indiquer quelles mesures concrètes seront prochainement adoptées pour gérer les détenus radicalisés et éviter que nos prisons ne soient davantage encore des lieux de radicalisation et d'apprentissage du terrorisme ?

syndicats. Ils ont quitté la table des discussions. Le Gouvernement en prend acte, mais appelle à la reprise du dialogue et au sens des responsabilités de chacun, car, comme vous le savez, la mission des personnels pénitentiaires ne peut pas être interrompue

Cette décision unilatérale, précipitée et prise sans concertation préalable avec les promoteurs du projet est une mauvaise nouvelle pour la France et pour la région capitale, dont je suis élue. Depuis le lancement officiel de l'association Expo France 2025, en 2013, lors d'une conférence au Grand Palais, à Paris, les soutiens politiques, les soutiens citoyens de tous bords sont venus renforcer cette formidable aventure collective. Cette décision est regrettable préjudiciable à la France, à plusieurs titres : un très grand nombre d'acteurs économiques étaient parties prenantes à ce projet, depuis la modeste PME jusqu'aux plus grands noms des réussites économiques de notre pays, et en permettaient le financement. l'Exposition universelle de 2025 aurait permis de mettre en valeur les savoir-faire et la capacité d'innovation de notre pays. En un mot, monsieur le Premier ministre, cela aurait contribué à son rayonnement.

Le 28 septembre dernier, nous avons franchi une étape supplémentaire avec le dépôt du dossier de candidature proprement dit. dit. À ce moment-là de la procédure, j'ai dit très clairement, très précisément, après m'être rapproché d'un certain nombre d'acteurs élus locaux, que l'État se réservait l'entière possibilité de ne pas donner suite à ce projet

18 janvier dernier, les deux personnalités chargées de l'analyse et de l'accompagnement du projet m'ont remis leur rapport.

que le modèle économique du projet comportait plusieurs faiblesses structurelles. En particulier, l'équilibre économique reposait, au moins à hauteur d'environ 300 millions d'euros, sur l'hypothèse d'une cession gratuite du foncier par l'établissement public d'aménagement Paris-Saclay. Or, une cession gratuite de foncier par un établissement public, c'est une subvention publique

ministre de l'intérieur. Madame la ministre, le Gouvernement a annoncé vouloir faire de la lutte contre les violences faites aux femmes une priorité. Je ne peux qu'approuver. Les violences au sein des couples, dont les femmes sont les premières victimes, comptent toutefois parmi les faits les plus difficiles à déceler. En France, tous les trois jours, une femme meurt sous les coups de son conjoint. À la Martinique, le dernier homicide perpétré dans le cadre conjugal date de ce week-end

En 2017, près d'un millier de plaintes concernant des faits de violences au sein du couple ont été traitées par les services de police et de gendarmerie martiniquais. Pour combattre un tel fléau, une seule arme : la connaissance. Aujourd'hui, Aujourd'hui, seulement un fait de violence conjugale sur dix est porté à la connaissance des services de police et de gendarmerie. Cette délinquance spécifique devrait être comptabilisée de manière distincte dans les statistiques.

de même pour les violences au sein du couple ? Un tel changement ne pourrait avoir que des vertus. Aussi j'attends une réponse positive de votre part ! La parole

Est-il nécessaire de préciser qu'il s'agit là d'une forte entrave au développement économique, à la création d'emplois, à la formation de nos jeunes et à la préservation de l'environnement ? Pourtant, une ligne ferrée existe. Reliant Carnoules, Brignoles et Gardanne, elle offre des possibilités de connexions vers Marseille et Nice. Cependant, elle est demeurée inutilisée durant des décennies, satisfaction de certains locaux, mais au plus grand détriment de nos concitoyens. Alors que les investissements dans notre réseau ferré ont concerné essentiellement les lignes à grande vitesse, pouvons-nous espérer du Gouvernement qu'il considère enfin que la priorité doit être désormais donnée aux transports locaux ?

par nos collègues du groupe interparlementaire d'amitié France-Madagascar et pays de l'océan Indien, que préside Mme Nassimah Dindar. La délégation vient de s'entretenir avec nos collègues Charles Guené,

La séance est reprise. Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social. Je rappelle que la discussion générale a été close. Nous passons à la discussion du texte

La généralisation de l'inversion de la hiérarchie des normes à l'ensemble du droit du travail a été engagée par la loi El Khomri, contre laquelle des millions de personnes s'étaient mobilisées. mobilisées. En effet, si le gouvernement précédent n'avait pas ouvert la boîte de Pandore de la libéralisation du droit du travail en inversant la hiérarchie des normes, en instaurant un barème indicatif des indemnités prud'homales en cas de licenciement abusif, en donnant une définition variable du licenciement économique selon la taille des entreprises et

Comme je l'ai dit en commission et lors de la discussion générale, cette tendance est ancienne. Elle suscite des craintes, mais je suis convaincu que nous devons accompagner cette réforme pour moderniser le code du travail et répondre aux attentes des partenaires sociaux dans les branches et dans les entreprises. Quel

contre laquelle des millions de personnes s'étaient mobilisées. Nous déplorons que le gouvernement précédent ait ouvert la boîte de Pandore de la libéralisation du droit du travail en promouvant cette évolution et en

des relations sociales dans la plupart des entreprises françaises et les discriminations subies par les représentants des salariés. En un sens, cette loi a dénaturé la finalité même du code du travail, lequel doit, d'abord, protéger le salarié dans le cadre du rapport de subordination qui le lie à son employeur, et non déterminer le niveau de flexibilité et de précarité de son contrat de travail.

continue d'exister dans le code du travail à travers la notion d'équivalence de garanties, utilisée pour autoriser un accord d'entreprise à traiter de sujets relevant normalement d'un accord de branche. L'avis de la commission est défavorable.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

L'article 1 ratifiant l'ordonnance relative au renforcement de la négociation collective réorganise les rapports entre la loi, les accords de branche et les accords d'entreprise. Au travers de cette ordonnance, le Gouvernement entend parachever l'inversion de la hiérarchie des normes en matière de droit du travail et la remise en cause du principe de faveur. Dans la continuité de la loi El Khomri, il s'agit d'élargir le champ de la négociation collective en généralisant la primauté de l'accord d'entreprise, ce qui contribuera à l'affaiblissement des protections légales et conventionnelles. Sur de nombreux points, le code du travail se trouve modifié dans un sens particulièrement régressif : primauté donnée à l'accord collectif sur le contrat de travail, instauration du référendum d'entreprise à l'initiative de l'employeur, élargissement des possibilités de négociation en l'absence de délégué syndical. Désormais, ce sont les accords d'entreprise qui fixeront les conditions d'emploi et de travail des salariés en matière de salaires minima, de classifications, de durée du travail, de droit à la formation, de mesures relatives aux CDD, aux CDI et aux nouveaux CDI dits « de chantier », d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, de mise à disposition de salariés temporaires auprès d'une entreprise utilisatrice, de rémunération des salariés portés, etc. Loin de simplifier le code du travail et de renforcer les droits des salariés, le texte entérine des reculs sociaux sans précédent. C'est pourquoi nous demandons la suppression de l'article 1er. La

l'avis de la commission ? Cette ordonnance comporte des apports importants sur des sujets aussi divers que l'articulation entre les accords de branche et les accords d'entreprise, l'instauration d'un régime juridique unique pour les accords de flexisécurité ou encore l'assouplissement des règles de mandatement syndical. Par ailleurs, cette réforme n'entraînera pas une concurrence sociale déloyale

Le scrutin est ouvert.

en réduisant les prérogatives des représentants syndicaux. Ainsi, il va être très compliqué, pour les syndicats, de diligenter une expertise pour faire annuler un plan social dont la mise en place entraînerait, par exemple, un risque avéré de surcharge de travail, comme ce fut le cas en 2013 à la FNAC. Pour prendre un exemple tiré de l'actualité, on imagine les conséquences redoutables qu'aurait l'application de ces ordonnances dans une grande entreprise comme Carrefour, dont la direction vient d'annoncer un plan massif de suppression d'emplois.

collectifs bénéficieront d'une présomption de conformité à la loi, et le licenciement d'un salarié qui refusera la modification de son contrat de travail sera réputé pour motif personnel et pour cause réelle et sérieuse. En d'autres termes, la signature du contrat de travail, tant par le salarié que par l'employeur, perd singulièrement de sa valeur. La question apparaît d'autant plus sérieuse lorsqu'on examine les conditions dans lesquelles les accords pourront

Elle permettra également aux employeurs des entreprises de moins de 50 salariés de négocier avec un salarié élu tout type d'accord. Cet amendement prévoit en complément les modalités de révision et de dénonciation de tels accords conclus dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, quel que soit leur effectif.

L'ordonnance rendra possible la négociation d'accords sans les syndicats dans les entreprises de moins de 50 salariés et permettra à l'employeur d'obtenir la validation d'un accord par référendum, en négligeant le rapport de sujétion inhérent à la relation de travail entre le chef d'entreprise et les salariés. Nous proposons donc de redonner leur place légitime aux syndicats dans les TPE, en supprimant le référendum et en restaurant le mandatement, dont nous pensons qu'il constitue une réponse adaptée dans les petites entreprises et qu'il permet le respect du droit des salariés.

parole est à M. Jean-Louis Tourenne. Nous proposons d'introduire la validation obligatoire de la commission de validation des accords collectifs pour les accords conclus par des élus non mandatés. Cela permettra de répondre à une double inquiétude quant au renforcement du rôle régulateur de la branche, d'une part, et à la remontée effective des informations de terrain au niveau de la branche,

dans les petites entreprises ne sont pas convaincantes. Les accords instituant les commissions paritaires régionales interprofessionnelles n'ont pas fait l'objet d'une évaluation loyale et sincère pour leur donner leur chance. L'amendement n° 80, présenté par MM. Tourenne

À défaut de salarié mandaté, nous ouvrons la possibilité de négocier à un ou des membres de la délégation du personnel du CSE. En outre, nous rétablissons l'obligation, pour l'employeur, d'informer les syndicats qu'il souhaite engager des négociations. M. Jean-Louis Tourenne. Les deux premiers paragraphes de l'article 8 de l'ordonnance n° 2017-1385 vont bien au-delà de ce qu'autorisait l'habilitation.

M. Guillaume Gontard. L'article 8 de l'ordonnance relative à la négociation collective prévoit que, dans les entreprises de moins de 11 salariés, l'employeur pourra, de manière unilatérale, soumettre à référendum ses décisions portant sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective. Le danger que présente cette mesure est flagrant : le référendum que vous voulez inscrire dans la loi n'est en aucun cas une forme de consultation démocratique. Les salariés seront en effet placés devant un choix binaire : accepter ou refuser les propositions qui leur sont soumises, sans pouvoir proposer une autre solution. Il existe évidemment un autre risque : que le refus soit immédiatement sanctionné, dans une forme de chantage à l'emploi tout à fait inacceptable. La logique référendaire est la négation même du dialogue social. C'est même la raison d'être de ce type de dispositif que de court-circuiter le dialogue social pour imposer la volonté patronale. C'est pourquoi nous proposons de supprimer cette prétendue nouvelle modalité de négociation et de lui substituer une procédure de mandatement dans les entreprises de moins de 50 salariés dépourvues de délégué syndical.

dans le code du travail des apports de la commission sur les règles de validité des accords collectifs signés par les élus du personnel dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, afin de tenir compte de la sixième ordonnance « travail

d'un délégué syndical. Comme on ne peut pas forcer un salarié à devenir délégué syndical, que le mandatement a montré depuis longtemps ses limites et que le n'est plus acceptable, il fallait bien proposer de nouvelles règles. Dans les entreprises de moins de 11 salariés dépourvues de délégué syndical, et dans celles qui emploient moins de 20 salariés et qui sont également dépourvues d'élus du personnel, l'employeur peut désormais conclure directement avec les salariés un accord collectif qu'il a préparé, portant sur l'un des thèmes ouverts à la négociation dans le code du travail, si les deux tiers du personnel l'acceptent. Dans les entreprises de 11 à 50 salariés dépourvues de délégué syndical, mais dotées d'élus du personnel, l'employeur qui souhaite conclure un accord a dorénavant le choix entre trois possibilités mises sur un pied d'égalité : il peut le signer soit avec des élus non mandatés, soit avec des élus mandatés, soit avec des salariés non élus, mais mandatés.

le Sénat, lors de l'examen de la loi Travail, avait déjà proposé une réforme similaire. La commission approuve donc cette réforme, qui permettra de développer de développer le dialogue social dans les petites entreprises, souvent oubliées du législateur, et qui pourrait susciter des vocations parmi les salariés pour rejoindre des syndicats, si ceux-ci changent leur stratégie et s'adaptent à cette nouvelle donne.

La commission est également défavorable à l'amendement n° 76, qui vise à redonner une forme de monopole aux élus mandatés pour conclure des accords dans les entreprises sans Nous avons tous constaté l'échec des règles antérieures. Aussi, nous devons essayer d'autres voies pour augmenter le nombre d'accords conclus dans les petites entreprises. L'amendement n° présenté par M. Tourenne, tend à introduire l'approbation obligatoire des projets d'accords négociés dans les entreprises dépourvues de délégué syndical par la commission paritaire de branche. L'obligation d'obtenir l'aval de la commission paritaire de branche serait, selon la commission, un frein

Cela dit, la proposition de notre collègue me semble intéressante et plus opérationnelle que le décret. J'avais proposé en commission un avis de sagesse, sous réserve

vote. J'ai entendu les explications fournies par Mme la ministre.

et auront pour mission de favoriser et d'encourager le dialogue social et la négociation collective dans les entreprises de moins de 50 salariés. Pour ce faire, il est prévu qu'ils établissent un bilan annuel du dialogue social dans le département, se prononcent sur toute difficulté rencontrée dans le cadre d'une négociation, sur la saisie d'un syndicat ou d'une organisation patronale, apportent leur concours ou leur expertise juridique aux entreprises dans le domaine du droit social. De plus, ils seront paritaires et à présidence tournante. En clair, ils risquent de ressembler à ces commissions régionales dont les représentants du patronat n'ont jamais accepté l'existence. On nous dira qu'il s'agit encore de réunions qui causent une perte de temps, alors que le vrai sujet- absolument insupportable -est que ces observatoires seront des tours de guet pour ce qui concerne la nature réelle du dialogue social dans les entreprises. De plus, ils pourront être saisis par un syndicat, et donc « mettre leur nez » dans cette demande au sein des petites entreprises, alors que chacun sait

En outre, leur utilité est douteuse, car leurs missions ne sont pas clairement identifiées et leurs prérogatives ne sont pas définies. Ces instances pourront être saisies par les partenaires sociaux de « toutes difficultés rencontrées dans le cadre d'une négociation », mais les services de l'inspection du travail, ainsi que la branche professionnelle, peuvent déjà jouer ce rôle de conseil juridique. Par ailleurs, le Sénat s'est toujours opposé à la multiplication des structures paritaires du dialogue social, comme les commissions paritaires régionales interprofessionnelles, les CPRI, qui méconnaissent la réalité du dialogue social dans les petites entreprises. Enfin, le Gouvernement, en publiant un décret dès le 28 novembre 2017 pour installer ces observatoires, avant même

Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable et que celui du Gouvernement est favorable. Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin est ouvert. Personne ne demande